L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le développement des plateformes numériques est aussi bien une source d'opportunités pour les travailleurs que de défis lancés à notre modèle social. Les travailleurs qui y recourent bénéficient d'une voie d'accès rapide à l'emploi, à l'emploi, le travail indépendant répondant aux aspirations du plus grand nombre d'entre eux. Pour autant, les plateformes n'ont pas toujours respecté le cadre permettant de garantir une indépendance réelle. C'est la raison pour laquelle le législateur a fait oeuvre de régulation à plusieurs reprises, pour corriger les écarts constatés entre le modèle du travail indépendant et la réalité des contraintes pesant sur les travailleurs. Notre conviction, c'est que nous devons tenir une position d'équilibre, qui permette à la fois d'accompagner le développement des plateformes de mise en relation et de mieux protéger les travailleurs qui y ont La voie que nous avons choisie est celle de la construction d'un dialogue social structuré et organisé entre les plateformes et leurs travailleurs, afin de bâtir des droits adaptés dans le cadre du travail indépendant. C'est tout le sens du projet de loi que Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports, et moi-même portons. Ce texte doit permettre de donner des droits sociaux aux travailleurs concernés. En réponse au développement des plateformes numériques, le principe de leur responsabilité sociale à l'égard de leurs travailleurs a déjà été progressivement affirmé.

En outre, les travailleurs ont acquis le droit de constituer une organisation syndicale et d'exercer un refus concerté de fournir leurs services sans être sanctionnés. La loi d'orientation des mobilités (LOM), que j'ai eu l'honneur de porter, a permis d'aller plus loin et d'instaurer de nouvelles garanties pour les travailleurs des plateformes de mobilité. À titre d'exemple, ces dernières doivent désormais communiquer, avant chaque proposition de prestation, la distance couverte et le prix minimal garanti de la course. Notre objectif est désormais d'aller plus loin que ce premier cadre et de donner un coup d'accélérateur au renforcement des droits des travailleurs. Tel est l'objet du présent projet de loi, qui doit permettre de structurer un dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité afin de mieux protéger les droits des travailleurs, sans remettre en cause les statuts existants. Vous le savez, ce gouvernement croit fermement dans les vertus de la démocratie sociale et dans la capacité des partenaires sociaux à concilier la protection des travailleurs et l'efficacité économique. La construction d'un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs doit faire émerger un socle de droits concertés et protecteurs. Il s'agit d'enrichir le droit du travail et d'y inclure l'ensemble des travailleurs, pour des raisons d'équité et de justice sociale. Nous sommes déterminés à permettre à ces travailleurs d'exercer leur activité dans des conditions dignes et suffisamment protectrices. cet égard, nous avons confié en janvier 2020 à Jean-Yves Frouin la mission de formuler des propositions sur la construction d'un tel dialogue social. Sur cette base, Bruno Mettling a ensuite bâti, dans la concertation, une feuille de route visant à structurer un tel dialogue pour les travailleurs des plateformes de mobilité. La première brique de ce dialogue social a été posée par l'ordonnance du 21 avril dernier, qu'il vous est proposé de ratifier dans le présent projet de loi. En votant ce texte, vous permettrez aux travailleurs des plateformes d'avoir accès à une représentation. Concrètement, pour chacun des deux secteurs d'activité concernés, celui des chauffeurs de VTC et et des livreurs à vélo, une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au début de l'année 2022. Cette élection permettra aux travailleurs indépendants d'élire les organisations qui les représenteront. Lors du premier scrutin, pourront être reconnues représentatives les organisations qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés. Les représentants désignés auront pour mission de construire des normes protectrices adaptées au secteur des plateformes. Ils bénéficieront de garanties particulières attachées à leur mandat, afin de les protéger contre tout risque de discrimination. La rupture du contrat liant l'un de ces représentants à une plateforme sera notamment soumise à autorisation administrative préalable. En parallèle, l'ordonnance du 21 avril 2021 prévoit la création de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), une instance qui permettra de faciliter le dialogue social. Cet établissement public aura pour mission de veiller au bon déroulement de l'organisation des élections professionnelles et de la mise en oeuvre des concertations. Le premier décret d'application de l'ordonnance a été publié mercredi dernier. D'autres le seront prochainement. La mission de préfiguration de l'ARPE prendra fin dans quelques jours, le nouvel établissement prenant ensuite le relais. C'est un pas historique que nous nous apprêtons à franchir : il permettra aux deux parties de mieux se comprendre et d'aboutir aux compromis nécessaires à une amélioration réelle et ambitieuse des droits. Grâce au texte que je vous appelle à voter largement, nous avançons sur la voie d'un socle de droits sociaux communs à l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. Si nous croyons aux effets positifs du dialogue social dans le cadre du salariat, il n'y a aucune raison de ne pas y recourir aussi pour consolider les droits sociaux des travailleurs des plateformes. Nous voulons toutefois aller plus loin encore pour finaliser le cadre législatif posé par l'ordonnance du 21 avril 2021, en vue de définir pleinement les modalités du futur dialogue social. Nous souhaitons aller au bout des préconisations de la mission coordonnée par Bruno Mettling

L'objectif de cet article est également de définir les règles relatives à l'organisation de la négociation collective, y compris les conditions de validité des accords, la définition de leur contenu, de leur format et de leur durée. Ces règles, que nous voulons fixer dans la loi, seront définies aussi bien au niveau du secteur d'activité qu'au sein des plateformes elles-mêmes,

permettre de fixer la liste des organisations représentatives des plateformes et de jouer un rôle de médiation en cas de différends entre les plateformes et les travailleurs. Par ailleurs, une habilitation est également prévue pour permettre au Gouvernement de renforcer les obligations applicables aux plateformes, afin de préserver l'autonomie des travailleurs indépendants. Nous souhaitons mieux informer les travailleurs lorsqu'ils reçoivent des propositions de prestation tout en préservant leur liberté de choisir et d'organiser leur activité. Je veux être très claire : le recours à ces ordonnances répond à un impératif d'efficacité, qui est de finaliser le cadre de ce dialogue social au printemps 2022, afin que les acteurs aient de la visibilité sur les règles applicables, car c'est à ce moment-là que seront organisées les premières élections des représentants des travailleurs des plateformes. répond aussi à un impératif méthodologique : celui de pouvoir consulter, dans le temps imparti, l'ensemble des parties prenantes, afin de déterminer avec elles les modalités adéquates que devra prévoir la loi.

Je me tiens d'ailleurs à la disposition des deux assemblées pour rendre compte devant elles de ces travaux avant la publication des ordonnances. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi doit nous permettre de franchir une étape décisive vers une meilleure protection sociale des travailleurs des plateformes. Son vote intervient moins de deux mois avant la présidence française de l'Union européenne, lors de laquelle nous défendrons l'idée d'une convergence sociale vers le haut en Europe. Nous avons l'occasion de tracer une voie équilibrée, ambitieuse et innovante, fidèle à notre histoire sociale. Ce texte nous permet de poser les premières briques d'un droit qui reconnaisse pleinement ces formes d'emploi, tout en offrant des protections à ces travailleurs. C'est par le dialogue social que nous pourrons bâtir une protection sociale nouvelle et équilibrée, qui réponde aux aspirations de près de 100 000 travailleurs indépendants. La parole

l'émergence ces dernières années des plateformes numériques de mise en relation a offert à de nombreux jeunes travailleurs sans formation, et parfois éloignés du marché du travail, l'opportunité d'exercer une activité professionnelle. Cette forme de travail indépendant doit ainsi être encouragée pour le potentiel d'emploi qu'elle représente. Mais cette forme d'activité peut aussi être porteuse de précarité sociale pour les travailleurs concernés. Leur relation contractuelle avec les plateformes est souvent déséquilibrée, en particulier dans les secteurs de la conduite de VTC et de la livraison. Cette précarité Cette précarité résulte également des lacunes de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui ne sont pas obligatoirement couverts en cas d'accident du travail et ne disposent pas d'une véritable assurance contre le risque de chômage. Les travailleurs des plateformes représentent encore une part modeste de l'ensemble des actifs. Toutefois, leur exposition médiatique a donné une acuité nouvelle à la question ancienne de la frontière entre salariat et travail indépendant. La Cour de cassation a parfois reconnu l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, mais sa jurisprudence n'est pas encore stabilisée. Dans son rapport de mai 2020 sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants, la commission des affaires sociales du Sénat estimait nécessaire de dépasser le débat sur le statut de ces travailleurs et de développer leurs droits de manière pragmatique, notamment par la voie du dialogue social. Le législateur a progressivement créé des droits spécifiques pour ces travailleurs indépendants, considérant que le salariat n'était ni souhaité par tous les travailleurs concernés ni compatible avec l'autonomie dont ils bénéficient pour exercer leur activité. La loi El Khomri du 8 août 2016 a ainsi posé le principe selon lequel les plateformes, lorsqu'elles déterminent les caractéristiques de la prestation et fixent son prix, ont une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs. Elle a également étendu aux travailleurs concernés certaines garanties fondamentales : une ébauche de droit de grève, ainsi que le droit de constituer une organisation syndicale. La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit des dispositions spécifiques aux secteurs des VTC et de la livraison telles que la possibilité pour les plateformes d'établir une charte de responsabilité sociale. Elle a par ailleurs prévu de nouveaux droits favorisant l'autonomie des travailleurs de ces secteurs. Ces dispositions sécurisent juridiquement le statut des travailleurs indépendants tout en répondant, en partie, à leur attente de protection.

Cette ordonnance prévoit que les travailleurs indépendants concernés pourront être représentés par des syndicats et des associations professionnelles, ce qui permettra d'intégrer celles qui oeuvrent déjà dans le champ des plateformes. La représentativité de ces organisations sera conditionnée au respect de plusieurs critères, dont le plus déterminant sera l'audience, laquelle sera mesurée par une élection. Les travailleurs des plateformes voteront pour les organisations candidates, sous réserve d'avoir une ancienneté de trois mois dans l'activité considérée. Les représentants désignés par les organisations déclarées représentatives bénéficieront de protections, de formation au dialogue social et d'indemnités pour l'exercice de leur mandat. Le premier scrutin devra se tenir avant la fin de l'année 2022 et sera organisé suivant des règles transitoires afin de faciliter l'émergence de premiers représentants des travailleurs. La commission a approuvé ces modalités de représentation, sous réserve que soient précisées les conditions pour être électeur, afin d'éviter que les travailleurs qui seraient électeurs dans les deux secteurs d'activité n'exercent deux fois leur droit de vote. Dans cette situation, le travailleur devra choisir le secteur dans lequel il votera. Bien entendu, ces dispositions ne constituent qu'une première étape dans l'élaboration d'un cadre permettant le développement du dialogue social. Elles s'inscrivent dans le contexte de travaux menés par la Commission européenne sur les possibilités de représentation collective et de dialogue social concernant des travailleurs indépendants et leur compatibilité avec le droit européen de la concurrence.

Cette mission, dont le coût est estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros par an, sera financée par une taxe acquittée par les opérateurs de plateformes. Cette autorité aura un rôle important de tiers de confiance à jouer dans la mise en place d'un dialogue formalisé entre les travailleurs et les plateformes. En revanche, la commission ne juge pas souhaitable que l'ARPE se mue en agence de régulation des secteurs économiques des plateformes de VTC et de livraison. Elle a donc précisé que l'objet de l'ARPE doit être circonscrit à la régulation du dialogue social entre les travailleurs et les plateformes des deux secteurs concernés. La commission a également supprimé la présence d'un député et d'un sénateur au conseil d'administration de l'ARPE, considérant qu'il n'est pas opportun de multiplier les organismes extérieurs au Parlement au sein desquels des parlementaires siègent ès qualités. Afin de compléter le cadre posé par l'ordonnance du 21 avril 2021, l'article 2 du projet de loi contient de nouvelles demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du texte. concerne la mise en place d'un dialogue social au niveau de chaque secteur d'activité, le Gouvernement serait habilité à prévoir par ordonnance les aspects qui n'étaient pas couverts par l'habilitation prévue par la LOM : les modalités de la représentation des plateformes, ainsi que les règles encadrant la négociation et le contenu des accords de secteur. Ce dialogue social sectoriel serait complété, à moyen terme, par l'organisation d'un dialogue social au niveau de chaque plateforme de mobilité. Un dernier volet vise à compléter par ordonnance les obligations incombant aux plateformes de mobilité afin de renforcer l'autonomie des travailleurs, de manière à sécuriser davantage la relation contractuelle entre les deux parties.

Les principaux enjeux du dialogue social en matière de régulation de l'économie des plateformes se situent au niveau sectoriel. La mise en place d'un dialogue social au niveau de chaque plateforme n'interviendra que dans un second temps. Dans cette perspective, le délai de douze mois prévu par le texte n'a pas paru approprié à la commission. Elle a donc supprimé tous les éléments de l'habilitation concernant l'organisation du dialogue social au niveau de la plateforme. Ce délai de douze mois paraît à l'inverse excessif pour la mise en place du seul dialogue social de secteur, alors que des travaux préparatoires ont largement tracé la voie à suivre au cours des deux dernières années. La commission a donc réduit à six mois la durée de l'ensemble de l'habilitation prévue à l'article 2. La commission a par ailleurs supprimé, par cohérence avec les modifications apportées à l'article 1, les alinéas visant à confier à l'ARPE, d'une part, un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs et, d'autre part, un rôle d'expertise, d'analyse et de proposition concernant l'activité des plateformes et de leurs travailleurs. Enfin, la commission a considéré que certains principes régissant la négociation de secteur devraient être débattus au Parlement et inscrits directement dans la loi. Elle a donc précisé, dans un nouvel article 3, que les organisations représentatives au niveau d'un secteur devront obligatoirement négocier, au moins tous les quatre ans, sur trois thèmes structurants communs aux deux secteurs la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels. Sous cette réserve, chaque secteur aura la possibilité de déterminer, pour ce qui le concerne, les domaines et la périodicité de la négociation collective. En effet, les travailleurs des deux secteurs concernés ont des aspirations différentes et ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. À défaut d'accord organisant le cadre de la négociation, les organisations devraient négocier chaque année sur la fixation du prix et tous les deux ans sur les autres thèmes obligatoires. Pour conclure, au-delà de la forme discutable de ce projet de loi, les dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2021 comme les orientations proposées à travers ces nouvelles demandes d'habilitation me semblent aller dans le bon sens. On peut toutefois regretter qu'elles ne concernent que les travailleurs de deux secteurs.

ces travailleurs restent donc très limitées, parallèles inquiétants de leurs conditions de travail. C'est une atteinte de plus à leur autonomie, mais plus grave encore, une atteinte à nos principes constitutionnels. En effet, ce texte porte atteinte aux principes fixés dans le préambule de la Constitution de 1946 relatifs au droit du travail et des salariés, ainsi qu'aux règles législatives du dialogue social, et ce pour trois raisons, madame la ministre. D'abord, le Gouvernement n'a pas respecté l'article L. 1 du code du travail, qui prévoit une concertation préalable obligatoire entre les organisations syndicales et patronales. Ensuite, le Gouvernement n'a pas respecté la décision du 26 janvier 2017 du Conseil constitutionnel, qui a rappelé que, aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, « le le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Enfin, le recours aux ordonnances sur les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes est contraire à l'esprit du Constituant de 1958 : le Gouvernement doit rattacher sa demande d'habilitation à l'exécution de son programme, au sens de l'article 49 de la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

leurs travailleurs, le Gouvernement a inscrit dans la LOM la possibilité pour les plateformes de rédiger, factuellement, mais toujours de manière unilatérale, des chartes relatives aux conditions de travail sans que ces textes puissent être invoqués devant les juges comme indices de subordination. disposition a été censurée partiellement par le Conseil constitutionnel au motif que le législateur avait ainsi permis aux plateformes de fixer des règles relevant de la loi.

La forme et le processus d'adoption amphigourique de cette ordonnance achèvent d'en faire la démonstration : c'est dans la LOM qu'avait été intégré un amendement permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnances pour organiser la représentation des travailleurs.

et moi-même avons menées dans le cadre de cette mission d'information ont pourtant permis d'identifier des solutions concrètes, comme le fait de consacrer dans la loi le principe d'une rémunération minimale pour les travailleurs, base sécurisante de négociation avec les plateformes. Et que dire des algorithmes,

organisent et contrôlent l'activité économique qu'elles ont créée, plaçant ainsi leurs travailleurs dans une dépendance économique. Il est donc fondamental que la négociation collective s'empare de ce sujet. Nous continuons de penser que, avec ce texte, vous tentez d'éviter l'inévitable, alors que la plateformisation de l'économie que vous défendez n'a jamais fait la preuve de sa rentabilité. Vous qui êtes si attachée à la liberté d'entreprendre et à l'autonomie des travailleurs indépendants,

jusqu'au principe même guidant la négociation collective. En effet, l'article 2 de la convention n° 154 de l'Organisation internationale du travail (OIT) définit la négociation collective comme s'appliquant à « toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur

du code du travail. Si l'on peut regretter le principe des ordonnances, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, il est tout à fait possible pour le Gouvernement de demander au Parlement une habilitation à prendre par ordonnance toute mesure relavant du domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel n'a jamais exigé que cette habilitation soit liée à une déclaration de politique générale. Enfin, ce projet de loi contribue à donner corps, pour les travailleurs concernés, à certains principes qui sont édictés par le préambule de la Constitution de 1946, notamment le droit pour tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Quel est l'avis du Gouvernement

permettant à ces acteurs d'engager des discussions sur le revenu minimal des travailleurs, la formation professionnelle ou la santé au travail. Plus vite seront fixées les règles permettant aux travailleurs de désigner leurs représentants, mais aussi de déterminer les thèmes de négociation, leur périodicité ou encore les règles de validité

Pour cela, le Gouvernement doit leur communiquer en amont « un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options Ce texte est de fait contraire à ces règles de la démocratie sociale. Même en l'absence de procédures de concertation, le Gouvernement, lorsqu'il décide de mettre en oeuvre un projet de réforme, doit faire connaître cette décision aux organisations en la motivant dans un document. Le projet de loi visant à créer ces organisations, celles-ci n'ont pu être sollicitées, par construction, ni être mises

il ne fait que refléter l'impact de la recherche d'un tiers-statut, qui fait l'unanimité contre lui - comme le rappelle la seconde motion, tendant à opposer la question préalable -et témoigne surtout de la volonté gouvernementale de sécuriser les plateformes contre le risque de requalification. le risque de requalification. Ce projet de loi, comme le relèvent d'ailleurs les deux motions, contrevient aux règles constitutionnelles qui imposent au Gouvernement de rattacher sa demande d'habilitation d'une ordonnance à l'exécution de son programme ou à sa déclaration de politique générale. Il illustre le bras de fer permanent engagé par le Gouvernement avec le Parlement. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe écologiste votera les deux motions. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

La parole est à Mme Monique Lubin, pour la motion. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le management algorithmique et l'économie de plateforme imposent leurs normes à la sphère du travail, rappelons les mots de Gilbert Simondon : « La machine peut se dérégler et présenter alors les caractéristiques de fonctionnement analogues à la conduite folle chez un être vivant. Mais elle ne peut se révolter. La révolte implique en effet une profonde transformation des conduites finalisées, et non un dérèglement de la conduite. La machine devenant le mètre étalon de l'évaluation de ce que devrait être le travail, le conformisme et la soumission menacent de s'ajouter à la recherche de l'efficacité à tout prix dans certaines sphères professionnelles. Dominique Méda a ainsi souligné, dans le cadre de la mission d'information du Sénat sur l'ubérisation de la société, que « le profil des livreurs a [ ...] changé. À l'étudiant s'est substitué le migrant sans papier, précaire et exploité. La plateforme donne certes de l'emploi, mais pour un travail de faible qualité. Il manque des cotisations sociales, alors que les plateformes sont des employeurs. On assiste à un contournement des obligations des employeurs, notamment pour le financement de la sécurité sociale ou des obligations de protection des employeurs Rappelons également que le fonctionnement de certaines applications pousse trop souvent les livreurs à jouer avec leur vie. Le statut des travailleurs de plateforme est le produit de l'exploitation des angles morts de notre système juridique par des agents économiques qui tendent à privatiser les bénéfices et à socialiser les pertes. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes ne menace pas d'y changer grand-chose. Il propose en effet la validation par le Parlement d'un dispositif de dialogue social mal ficelé, et renvoie - une fois encore - à des ordonnances ! Loin de conforter la démocratie d'entreprise, il menace de susciter une pratique exotique, un dialogue social organisé autour de syndicats d'indépendants, ce que l'on pourrait appeler un cartel, ou une entente. La place centrale de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) dans ce dispositif pose aussi question. Loin d'avoir une vision de ce que doit être le travail dans le cadre de l'économie numérisée, ce qui aurait légitimé un projet de loi ambitieux, le Gouvernement adopte une stratégie du bricolage pour banaliser un état de fait. Le texte que nous examinons aujourd'hui participe en effet de la constitution à bas bruit d'un tiers-statut pour les travailleurs de plateformes. Cette tactique des petits pas permet au Gouvernement de dissimuler ce qu'il est en train de faire, et qu'il se garde bien de nommer ou de revendiquer. La mise en oeuvre de cette tactique s'accélère. Le Gouvernement ne cesse de faire légiférer en ce sens, aussi bien implicitement qu'explicitement. La constitution de ce tiers-statut est d'abord bien sûr explicite dans le cadre du présent projet de loi, discuté dès juillet 2021 à l'Assemblée nationale. Dans le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante débattu au mois d'octobre 2021, le sujet des travailleurs de plateforme n'est par ailleurs abordé à aucun moment. Cela aurait pourtant été l'occasion de clarifier leur statut, puisqu'ils sont supposés être des travailleurs indépendants ! La tâche aurait certes été difficile, car, comme nous le savons, une partie écrasante d'entre eux est économiquement dépendante. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, un amendement du Gouvernement a créé l'article 50 , qui a pour objet de faire bénéficier les travailleurs des plateformes du régime général de la sécurité sociale sous réserve d'un revenu annuel inférieur à 1 500 euros.

La majorité du Sénat semble entériner la démarche de l'exécutif, puisqu'elle a fait le choix de compléter le présent projet de loi, dans un double mouvement. Elle prétend d'une part vouloir contrôler les excès politiques du texte par la suppression d'une ordonnance, la réduction à six mois de la validité d'une autre, et le refus que les parlementaires siègent à l'ARPE. Dans le même temps, elle apporte sa pierre à l'édifice en encadrant le dialogue social proposé par le Gouvernement. Comme la majorité du Sénat, le Gouvernement fait le choix d'aller à rebours du sens de l'Histoire, celui d'une modernité démocratique qui marque pourtant des points à travers le monde. Des activistes, des professionnels, des acteurs politiques, juridiques et syndicaux réussissent à renverser la vapeur face au rouleau compresseur de l'ubérisation. Nous avons tous en tête les décisions prises au Portugal, où les plateformes de commande de repas en ligne telles qu'Uber Eats et Glovo sont obligées de proposer à certains de leurs livreurs des contrats et des avantages formels. En Espagne, la loi , adoptée mi-mai par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, a permis ces dernières semaines l'embauche de milliers de coursiers jusqu'alors considérés comme indépendants. détaillerai pas ce qui se passe en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, en Californie ... Je rappellerai, en revanche, les décisions des instances juridiques françaises, cours d'appel et Cour de cassation, qui ont fait mouvement vers la requalification salariale. La multiplication des coopératives de livraison fait par ailleurs la démonstration du refus des professionnels de se soumettre à un modèle qui ne leur convient pas. Il y a enfin la résolution du Parlement européen, en date de septembre 2021, qui acte tout à la fois qu'un tiers-statut n'est pas souhaitable, qu'il conviendrait de classer les travailleurs de plateforme soit comme de véritables indépendants, soit comme des salariés, et qui promeut une présomption réfragable de relation de travail.

Madame la ministre, vous avez explicité votre position auprès de notre collègue député Boris Vallaud lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Vous avez déclaré souhaiter « la poursuite d'une activité économique créatrice d'emplois, qui peut par ailleurs permettre une insertion professionnelle rapide pour un certain nombre de travailleurs, tout en garantissant un socle de droits sociaux ». C'est dire l'ambition de votre gouvernement donner des privilèges exorbitants à des plateformes, ce qui passe par l'extrême fragilisation de notre modèle social, en échange d'un droit de survie pour des travailleurs économiquement dépendants, qualifiés d'indépendants et victimes d'un tiers-statut. autre point a été explicité au cours des débats à l'Assemblée nationale : le fait que les dispositions du présent projet de loi vous donnent l'opportunité d'effacer les liens de subordination entre les plateformes et les travailleurs, alors qu'elles sont l'élément clef d'une possibilité de requalification salariale que nous appelons de nos voeux au profit des travailleurs qui le souhaitent. approche tactique, qui procède par bricolages successifs pour aboutir à la validation d'un état de fait imposé par les plateformes, est nocive à court, moyen et long terme. Le rejet unanime du tiers-statut emprunte de fait ses arguments du côté de l'insécurité juridique qu'il introduirait pour les entreprises. C'est ce que mettent notamment en avant le rapport Frouin et la résolution du Parlement européen de septembre dernier. Le soutien aux indépendants est antinomique de la création de ce tiers-statut : si les professionnels indépendants doivent travailler avec les plateformes, il faut que cela soit dans des conditions respectueuses de ce statut. De fait, le tiers-statut créerait, comme le souligne également la résolution du Parlement européen, une situation de concurrence difficilement supportable pour ces derniers. Fragilisant le statut salarial aussi bien que le statut des indépendants, le tiers-statut que le Gouvernement est en train de mettre en place est un véritable trou noir, susceptible de vider de leur substance salariat et indépendance. Et les menaces qu'il fait peser sur notre modèle social sont d'une gravité sans précédent. Au sein de cette enceinte parlementaire, nous avons lutté contre cette approche choisie par le Gouvernement. Nous avons bataillé, en juin 2018, dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, puis en novembre 2018 au cours de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, contre la volonté du Gouvernement d'offrir aux plateformes le moyen de se dédouaner de leurs responsabilités sociales - notre recours au Conseil constitutionnel sur le sujet ayant d'ailleurs connu le succès que l'on sait.

Le recours aux coopératives, dont nous avons souligné l'intérêt, est également identifié comme une piste à explorer dans le rapport Frouin ou dans la résolution du Parlement européen. La proposition de loi contre l'indépendance fictive des travailleurs des plateformes, débattue en mai dernier et portée par Olivier Jacquin, moi-même et le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, proposait quant à elle de nombreuses solutions dont l'intérêt saute aux yeux une procédure de requalification par action de groupe ; la suppression de la présomption de non-salariat et son remplacement par une présomption de contrat de travail ; la possibilité pour les conseils de prud'hommes saisis de demandes de requalification d'exiger la production de l'algorithme utilisé par une plateforme et celle de recourir, si nécessaire, à un expert. Alors que se profile le métavers, où la frontière entre le réel et le virtuel menace de se brouiller jusqu'à disparaître complètement, et qui est un projet d'altération du monde du travail bien plus massive que celle causée aujourd'hui par les plateformes numériques, le Gouvernement ne semble pas avoir saisi l'ampleur de sa responsabilité, historique, de fixer un cadre et des règles au monde du travail qui soient conformes au modèle social et politique que nous nous sommes choisi. Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estime pour sa part qu'il n'est pas possible de légiférer en catimini et de procéder par glissements successifs sur un enjeu majeur pour notre modèle social. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de présenter devant notre assemblée cette motion tendant à opposer la question préalable.

pour bâtir des droits adaptés dans le cadre du travail indépendant, tout en respectant les statuts existants. Nous entendons aussi respecter la volonté des travailleurs, dont une majorité écrasante souhaite une amélioration de leurs droits, tout en préservant leur statut d'indépendant, qui leur procure souvent une autonomie et une liberté d'organisation à laquelle ils sont attachés. Je crois en la capacité du dialogue social à tirer vers le haut les droits des travailleurs. Je crois en la responsabilité des acteurs pour définir un cadre mieux-disant, tant au bénéfice des travailleurs que des plateformes elles-mêmes, qui ont là un véritable enjeu d'attractivité et de réputation. Pour autant, nous devons structurer ce dialogue social et le rendre exigeant pour permettre aux travailleurs concernés de définir les solutions les plus adaptées à un environnement de travail très spécifique et en pleine mutation. Je voudrais être claire : ces ordonnances n'enlèvent n'enlèvent rien au pouvoir du juge de requalifier en salarié un travailleur qui ne serait pas réellement indépendant. Il ne s'agit pas de réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination entre une plateforme et ces travailleurs.

dans le cadre de ce dialogue social. Si vous adoptez cette habilitation, le Gouvernement reviendra naturellement devant vous avec un nouveau projet de loi de ratification de l'ordonnance à l'issue du délai imparti par l'habilitation. Le Parlement sera donc de nouveau associé pleinement à l'écriture des modalités du dialogue social, comme aujourd'hui.

Comment pouvez-vous nous dire que cela ne vise pas à enlever des possibilités de requalification au juge ? Dans l'étude d'impact, clairement, on parle de sécuriser juridiquement le modèle économique des Je citerai tout à l'heure la rapporteure du texte pour l'Assemblée nationale, qui a été d'une transparence éloquente. Elle a clairement dit qu'il s'agissait précisément de réduire le faisceau d'indices - vous ne l'avez pas contredite à

Mais nos acteurs économiques, petits patrons, commerçants, artisans ont sacrément d'autres contraintes que les plateformes numériques de travail !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de saluer notre rapporteur, Mme Frédérique Puissat, pour la clarté de son rapport et l'esprit de lucidité qui en émane. Madame la ministre, Madame la ministre, à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que l'on ne pouvait s'opposer à ce texte, « ni par idéologie ni par principe. » Mais l'idéologie et les principes sont derrière chaque choix politique et économique ! La sécurité sociale, les congés payés ont été d'abord des principes avant d'être reconnus, plus tard, comme des choix politiques considérés comme relevant du pragmatisme. La dignité, l'épanouissement au travail et par le travail nécessitent de faire appel à de profondes convictions. Les travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, souvent par la microentreprise, comme principale activité ou comme complément d'activité, adhèrent, plus ou moins consciemment, à une forme de travail porteuse de précarité sociale. Cette précarité repose sur un principe simple : un déséquilibre de la relation contractuelle entre le travailleur indépendant et la plateforme. Derrière ce modèle, accepté autant par les travailleurs indépendants que par certains consommateurs, il y a le choix du moindre mal, c'est-à-dire : tout plutôt que le chômage. Ce choix mérite d'être reconnu, accompagné, voire valorisé, mais ne pourrions-nous pas, madame la ministre, identifier ces travailleurs et reconnaître leur bonne volonté en leur proposant davantage de formations, ou tout autre type d'accompagnement qui leur serait bénéfique ? Comment ne pas être convaincu par le fait que le modèle économique des plateformes aura permis, comme le souligne Frédérique Puissat, un recours plus facile à l'emploi ? Les plateformes auront offert à de nombreux jeunes travailleurs sans formation, et parfois éloignés du marché du travail, l'opportunité d'exercer une activité professionnelle. Tout laisse à croire que ce modèle économique s'étendra à d'autres secteurs d'activité. En 2008, le secrétaire d'État Hervé Novelli indiquait : « Quel meilleur ascenseur social que l'autoentreprise ? Elle ne nécessite ni moyens, ni diplômes, ni relations. » Seulement, au-delà de la belle aventure entrepreneuriale, le Président de la République, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, faisait le triste aveu suivant : «

la lutte contre le chômage doit passer par le dumping social au détriment de la prévention, de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs, les Français auront du souci à se faire. L'injonction consistant à limiter les droits au nom de la lutte contre le chômage a évidemment ses limites. Il n'a pas fallu attendre quatre ans après l'apparition d'Uber en France, en 2012, pour que la loi appelle à la « responsabilité sociale » des plateformes, permettant la prise en charge, directe ou indirecte, d'une assurance couvrant le risque d'accident du travail ou la contribution à la formation professionnelle. En 2018 et en 2020, la Cour de cassation a reconnu à un livreur, puis à un chauffeur de plateforme le statut de salarié. Ces deux arrêts majeurs constatent le pouvoir de contrôle et de sanction reconnu aux plateformes, pouvoir » qui qualifie en droit la relation de subordination salariale. Ils font écho à des décisions de requalification prises dans d'autres États, de la Californie, où est né Uber, à l'Italie, en passant par le Royaume-Uni. Car oui, rappelons-le, des pays plus libéraux que le nôtre, comme les Pays-Bas ou la Suisse, sont allés plus loin dans la protection des travailleurs indépendants des plateformes. Nous vous encourageons à poursuivre l'effort. avec ce projet de loi, qui pose les bases d'un dialogue social structuré entre plateformes et travailleurs indépendants, vous ajoutez une pierre à l'édifice. L'ordonnance permet notamment d'accompagner le dialogue social, d'organiser les élections professionnelles, d'établir les listes électorales, de financer la formation des représentants et de promouvoir le dialogue social. Nous saluons cette avancée, même si nous aurions espéré que l'ordonnance soit étendue à d'autres secteurs. La création de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), chargée de réguler le dialogue social entre travailleurs indépendants et plateformes, permettra, nous l'espérons, aux indépendants de défendre un statut auxquels ils sont attachés et d'acquérir des droits nouveaux en matière de protection sociale. Pour autant, nous le savons, les conditions du dialogue social et des négociations sont le corollaire d'un rapport de force qui n'est pas favorable aux travailleurs indépendants. Cela nous permet de comprendre pourquoi les plateformes saluent votre ordonnance. Il est par conséquent important de garantir un dialogue social équilibré et de donner corps à ces négociations. Cela passera par la définition d'un socle restreint de thèmes de négociations

Le présent projet de loi est discutable sur la forme et incomplet sur le fond. Les orientations envisagées dans les dispositions de l'ordonnance, mieux encadrées par notre commission des affaires sociales, semblent aller dans le bon sens.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, je souligne l'urgence pour le législateur de réguler des questions ayant trait à la numérisation de notre société, tant celle-ci subit des transformations majeures à un rythme de plus en plus rapide. Il relève ainsi de l'évidence que l'importance croissante des plateformes numériques participe à une modification substantielle de la structure de notre économie, qu'il s'agisse de la communication, de la consommation ou du travail. Et c'est bien là toute la légitimité de l'intervention du législateur, dans la mesure où les droits des travailleurs ne peuvent pas rester à la traîne des mutations systémiques de l'économie. De nombreuses questions se posent donc en filigrane. Comment garantir une protection sociale optimale à ces travailleurs que le droit a du mal à qualifier ? Comment appréhender la nature de la relation contractuelle entre les plateformes et ces travailleurs ? Comment mettre en place les conditions d'un réel dialogue social lorsqu'émerge un nouveau secteur ? ? Dans ce contexte, le texte que nous examinons aujourd'hui vise à autoriser la ratification d'une ordonnance relative au dialogue social entre les plateformes numériques et les travailleurs qui y ont recours. Pour rappel, le processus de régulation des plateformes a débuté en 2016 avec la loi El Khomri, qui consacre leur responsabilité sociale. Depuis lors, ces dernières prennent en charge les assurances couvrant les risques d'accidents du travail ou encore participent financièrement aux formations des travailleurs indépendants.

de la définition des règles de représentativité des plateformes ou encore de l'introduction d'une obligation de formation et de consultation des plateformes au bénéfice des travailleurs qui y recourent. Malgré leur statut en marge des catégories classiques du droit du travail, ces travailleurs vont donc bénéficier de règles tendant vers le droit commun. En somme, mes chers collègues, le texte viserait à restructurer favorablement l'asymétrie qui caractérise la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants. Bien que l'intention de lutte contre la fragilité et la précarité des travailleurs indépendants concernés semble claire, je m'interroge sur l'efficacité du dispositif à l'étude. Madame la ministre, votre projet de loi décompose temporellement en deux parties le dialogue social ; d'abord sectoriel,

Ne risque-t-on pas de miter les avancées sociales promises par ce texte ? N'oublions pas que le législateur doit permettre le développement des plateformes en garantissant l'évolution des droits sociaux de tous les travailleurs, sans distinction. Si la loi est la même pour tous, les droits des travailleurs indépendants doivent être les mêmes. Notre groupe tient également à rappeler l'importance de l'intégration des partenaires sociaux dans tout type de négociations. Nous appelons le Gouvernement à être attentif à leur juste mise en relation avec l'ARPE. Quoi qu'il en soit, l'objectif de Quoi qu'il en soit, l'objectif de régulation du texte reste compréhensible et permet d'avancer relativement dans la construction du dialogue social. Dommage qu'il s'effectue par ordonnance. Cette procédure ne peut remplacer le nécessaire travail parlementaire et les solutions plus rassurantes et étayées qui auraient pu être

LOM en 2019. Je ne pourrai donner la position de mon groupe sur ce texte sans avoir préalablement mis en évidence le piège qui nous est tendu : cette construction par ordonnances croisées vise à créer un tiers-statut, alors que l'on prétend l'inverse indiquant vouloir améliorer la situation de travailleurs précaires par le dialogue social. Madame la ministre, n'êtes-vous pas étonnée que, dans les deux assemblés,

cela ne tient pas seulement au fait que, tout en prétendant vous faire le chantre du dialogue social, vous écrasez une nouvelle fois le Parlement par une double ordonnance. Je ne sais d'ailleurs

Le rapport de Pascal Savoldelli, intitulé, adopté à l'unanimité, a clairement mis en évidence que le secteur des livreurs et VTC était l'arbre qui cachait la forêt. La gangrène de la plateformisation du travail s'étend à de nombreux secteurs du fait du dévoiement du statut d'autoentrepreneur. Il est urgent de la contrôler à travers une puissante autorité indépendante, pas cette ARPE, dont les faibles attributions

Alors que nous dressons tous peu ou prou les mêmes constats sur les dérives de la plateformisation, je reviens sur vos intentions. Elles ont été parfaitement révélées par la rapporteure du texte

est de « réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination, tel que celui-ci est défini par la jurisprudence, entre les plateformes et les travailleurs,

il est- je pèse mes mots - perfide de qualifier de « dialogue social » l'octroi de quelques menus droits aux indépendants fictifs pour s'assurer qu'ils ne puissent pas être requalifiés.

Madame la ministre, quand la Cour de cassation, le 4 mars 2020, puis la cour d'appel de Paris, le 16 septembre 2021, parlent d'indépendance fictive, donc d'illégalité, vous y voyez y voyez un « risque pour le modèle économique des plateformes ». Vous continuez de vouloir plus protéger les plateformes que les travailleurs qu'elles emploient.

Ce texte permet de sortir de l'ambiguïté. Ceux qui le voteront ne pourront plus dire qu'ils n'en voulaient pas ! À ce sujet,

Vous paraissez à moitié consentante, convertie au « en même temps ». Je vous le dis : vous y êtes favorable, et vous allez le révéler par votre vote

qui s'affranchissent de nos règles et s'exonèrent du code du travail ? Quelle distorsion de concurrence, pourtant ! Que faites-vous pour assurer une égalité de traitement entre les petites entreprises, qui payent leurs cotisations à l'Urssaf et se font contrôler régulièrement par l'inspection du travail, et les plateformes, qui Et que faites-vous concrètement pour lutter contre le travail dissimulé, qui ne se cache même plus avec le développement des sous-locations de comptes en cascade ? Vous ne faites pas respecter le droit du travail ! Pire, vous venez nous parler de dialogue social dans ces conditions

En effet, les travailleurs auraient dû élire des représentants sans connaître l'objet et le contenu des futurs accords qu'ils auront à négocier. Vous leur promettez donc à présent qu'ils pourront discuter, notamment, des rémunérations. que ces travailleurs sont des indépendants, vous confirmez qu'ils sont juridiquement des entreprises. Comment, dès lors, les autoriser à se regrouper pour aller négocier ? À l'instar du Conseil d'État, qui évoque une « applicabilité incertaine », nous contestons la conformité de cette disposition avec le droit de la concurrence, notamment régi par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tant que ce droit n'a pas bougé. Mais d'autres interrogations demeurent. Qu'en est-il concrètement des conditions de représentation des plateformes ? Seront-elles représentatives selon leur chiffre d'affaires, comme vous l'avez évoqué à l'Assemblée nationale ? Cela me semblerait un dispositif étonnant. Y aura-t-il une pondération selon le nombre de travailleurs inscrits ? Il y a des dizaines de critères qui méritent un vrai débat parlementaire. Et je ne parle même pas des travailleurs qui se feraient déconnecter quelques jours avant les votes, de sorte que l'audience des plus influents soit réduite Chers collègues, ne faites pas le choix de la précarité contre un peu d'activité, car d'autres modèles existent. Regardez les plateformes Take Eat Easy ou Gorillas, qui embauchent en parce que le modèle de livraison avec des autoentrepreneurs est dévoyé et dégradé. Regardez l'Espagne, qui a mis en place la présomption de salariat, solution que nous, sénateurs socialistes, proposition de loi rejetée au mois de mai. Mais surtout, regardez le Parlement européen, qui reprend également dans sa résolution du 16 septembre la présomption de salariat et l'inversion de la charge de la preuve en matière de requalification. Ce rapport a été remis par Sylvie Brunet, députée européenne En Marche, et voté par une très large majorité, dont une bonne partie des je me réjouis d'entendre que le commissaire européen Nicolas Schmit devrait reprendre les grandes orientations de cette résolution dans le projet de directive sur les travailleurs des plateformes qu'il présentera le 8 décembre.

dangereux pour notre modèle social, dangereux pour la valeur travail, qu'il abaisse, dangereux par les distorsions qu'il crée dans l'économie. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cheval de Troie contre nos valeurs de solidarité et de justice.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, c'est un rendez-vous presque régulier : ces derniers mois, nous avons en effet eu l'occasion de débattre ici de plusieurs propositions de loi relatives aux conditions de travail et à la représentation des travailleurs indépendants des plateformes. La dernière d'entre elles, déposée sur l'initiative de nos collègues socialistes, prévoyait- c'était au mois de mai dernier -d'étendre les actions de groupe aux procédures de requalification et de supprimer la présomption de non-salariat en cas de management algorithmique. Nous nous étions opposés à de telles dispositions au motif qu'en ce qui concerne les actions de groupe, il existait autant de cas de figure que de plateformes et de travailleurs et qu'une solution unique ne nous semblait pas adéquate. Nous avions également avancé que les décisions des différentes cours d'appel et des conseils de prud'hommes avaient démontré que le droit existant répondait déjà en partie aux attentes des travailleurs, puisqu'il assure la prise en compte du caractère unique de chaque situation. Il nous semblait enfin abusif de considérer que la requalification des travailleurs était une demande pleinement partagée. Il apparaît en effet clairement qu'une majorité des travailleurs indépendants souhaitent souhaitent conserver l'agilité que leur permet ce statut, motif pour lequel nous avions également souhaité conserver la présomption de non-salariat. Pourtant, la méthode qui était alors proposée, il nous apparaît urgent de faire évoluer le cadre juridique qui gouverne les relations professionnelles entre les plateformes et les travailleurs indépendants, en particulier dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur et celui de la livraison. Le développement exponentiel de ces plateformes et du nombre de travailleurs qui y ont recours appelle en effet une réponse rapide de la part du législateur et un dialogue social renforcé, seul à même, selon nous, d'assurer aux travailleurs des plateformes numériques les droits et la souplesse que leur statut d'indépendant leur garantit.

par voie d'ordonnance les modalités de représentation des travailleurs indépendants. C'est cette nouvelle ordonnance du 21 avril 2021 qu'il nous est proposé aujourd'hui de ratifier. L'article 1 du projet de loi prévoit ainsi la création de trois nouveaux chapitres au sein du code du travail. Il instaure un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs qui les utilisent au sein de deux secteurs d'activité : les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) et les activités de livraison. Il crée par ailleurs l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de réguler les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs indépendants. L'article 2 prévoit l'habilitation du Gouvernement à prendre des mesures par voie d'ordonnance, afin de préciser la structuration du dialogue social entre les plateformes numériques de mobilité et les travailleurs indépendants, avec pour objectif de finaliser le cadre d'un nouveau dialogue social dans les mois à venir. En commission des affaires sociales, le Sénat est revenu sur plusieurs dispositions d'un texte que nous pensions pourtant équilibré. Il a adopté la réduction de douze à six mois de l'habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social des plateformes.

La majorité sénatoriale a, par voie de conséquence, souhaité inscrire directement dans le projet de loi les domaines et la périodicité de la négociation collective au niveau de chacun des secteurs d'activité concernés par la mise en place d'un dialogue social. Nous regrettons ces modifications, qui, dans les faits, retarderont en plus de contraindre la structuration du dialogue social entre les plateformes numériques et les travailleurs indépendants qui y ont recours, et ce alors même nous, le temps est compté. Nous regrettons également la suppression du rôle de médiateur de l'ARPE, suppression qui laisse un vide, si ce n'est un flou, que la nouvelle rédaction ne nous semble pas combler. Les missions de médiation et d'expertise de l'ARPE nous apparaissent en effet particulièrement utiles pour accompagner la mise en place d'un dialogue social équilibré et constructif, capable de garantir agilité et protection. J'ajouterai qu'il est crucial de finaliser le cadre de ce dialogue social avant le début de l'année 2022, afin que les premières élections des représentants des travailleurs des plateformes puissent avoir lieu. C'est pourquoi notre groupe votera les amendements de rétablissement déposés par le Gouvernement. Il se prononcera en faveur de ce projet de loi de ratification et d'habilitation, qui, malgré les modifications apportées par le Sénat, demeure

La crise sanitaire a été un accélérateur, notamment durant les périodes de confinement. Elle a entraîné le développement des applications de livraison alimentaire en deux-roues. La livraison de commandes à domicile constitue un nouveau mode de consommation. Il en est de même pour le transport, avec l'explosion du recours aux VTC dans les grandes villes. L'arrivée de ces plateformes est ainsi venue remettre en cause nos conceptions classiques du travail. En effet, l'essor de ces nouveaux services a quelque peu dérouté les gouvernants et le législateur, car aucun texte ne prévoyait d'encadrement juridique et social

D'ailleurs, à un moment où notre pays est confronté à des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs et où il y a des débats sur la conception et la valeur du travail, nous pouvons noter que malgré une protection sociale quasi inexistante, des salaires peu élevés et des horaires compliqués, le secteur se développe et crée de l'activité.

par la prise en charge d'une assurance couvrant le risque d'accident du travail et de la contribution à la formation professionnelle ou des frais d'accompagnement des actions de formation permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Il a également été reconnu à ces travailleurs le droit de constituer en organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leur intérêt collectif. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 2019 a établi une charte déterminant les droits et obligations des plateformes, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Et elle a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures concernant les modalités de représentation des travailleurs indépendants et les conditions d'exercice de cette représentation.

travailleurs indépendants. Si l'émergence et le développement de nouvelles formes de travail ouvrent des perspectives économiques nouvelles, ils engendrent également des défis sociaux nouveaux. Cela nécessite une adaptation de notre droit, afin de garantir un dialogue social équilibré.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe partage le constat effectué par notre rapporteur : le développement rapide des plateformes répond à la fois à une demande des utilisateurs et au souhait d'indépendance exprimé par certains actifs, qui peuvent ainsi éviter la subordination et les contraintes liées au statut de salarié. Il permet également à des travailleurs peu qualifiés d'exercer une activité. Mais ces travailleurs ne sont ni tout à fait des travailleurs indépendants, compte tenu de l'absence de liberté dont ils disposent généralement dans l'exécution de la prestation ou dans la fixation de son prix, ni vraiment des salariés,

Dépasser la question du statut pour développer le dialogue social entre travailleurs et plateformes permettrait, en effet, de répondre de manière pragmatique au besoin immédiat de protection sociale de ces travailleurs. Nous nous réjouissons que le présent texte vienne concrétiser ces propositions, même si nous regrettons que le calendrier retenu par le Gouvernement interfère avec les travaux menés au niveau européen, pour s'inscrire dans la période préélectorale. Sur la forme, nous sommes opposés au recours aux ordonnances, qui dessaisit le Parlement de ses compétences. L'article 1 ne soulève pas de difficultés, car il prévoit la ratification de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative à la représentation des travailleurs, dont nous connaissons et approuvons le contenu. Le champ de l'habilitation prévu à l'article 2 est, en revanche, beaucoup plus large et indéterminé. Des amendements adoptés en commission ont permis de l'encadrer strictement. Nous pouvons donc approuver son contenu resserré. Conformément à la LOM, ce projet de loi représente une première étape consistant à organiser un dialogue social dans les deux secteurs de la conduite de VTC et de la livraison en véhicule, les travailleurs en relation avec des plateformes y étant exposés à des risques particuliers et à une certaine précarité. Le rapport sénatorial de mai 2020 proposait le choix de thèmes de négociation obligatoires, tels que la fixation du tarif, le développement des compétences et la prévention des risques professionnels. Je tiens ici à saluer la qualité du travail de notre rapporteur, qui a complété le projet de loi, en introduisant ces thèmes dans un nouvel article 3 adopté en commission. Cette disposition, une fois inscrite dans la loi, assurera une négociation tous les quatre ans, voire de façon plus rapprochée, à défaut d'accord encadrant la négociation. Nous ne suivrons pas le Gouvernement dans sa volonté d'organiser un dialogue social au niveau de chaque plateforme- ce qui est prématuré -ni dans son souhait de rétablir le champ de son habilitation, qui visait des aspects non mentionnés par la loi LOM et dessaisissait le Parlement. Nous nous opposons également à la réintroduction d'amendements qui tendraient à faire de l'ARPE une agence de régulation des secteurs économiques des plateformes de VTC et de livraison.

pour la durée de l'ensemble de l'habilitation prévue à l'article 2. L'étape fondamentale que nous franchissons aujourd'hui repose sur le poids donné à la négociation collective.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons peut, à certains égards, apparaître comme un progrès pour les travailleurs des plateformes.

Certes, les travailleurs disposent désormais d'un cadre régissant le dialogue social. Pour autant, ils n'ont toujours pas de salaire minimum, toujours pas de protection contre les licenciements par déconnexion de la plateforme, toujours pas d'encadrement de la durée maximale de travail, toujours pas de congés ni de jours de repos garantis et rémunérés. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à ratifier une ordonnance volontairement vide, puisqu'elle renvoie les conditions de travail à la négociation collective, sans protéger les travailleurs ni corriger, surtout, les inégalités de rapport de force entre les plateformes et les travailleurs. Sans institutions publiques et juridiques protectrices, rien ne contrebalance le poids prépondérant des plateformes face à leurs subordonnés. J'utilise ici à dessein

La véritable raison pour laquelle les plateformes ne veulent pas entendre parler de salariat réside dans leur modèle économique, dont les fondements reposent non pas sur la rentabilité économique, mais sur les mannes de fonds d'investissement qui leur permettent de croître rapidement, d'entrer en bourse, de capitaliser sur leur valeur boursière et de distribuer des dividendes.

matière, la variable d'ajustement est toujours le travailleur, qui voit le tarif de ses prestations fluctuer selon le bon vouloir des plateformes, et qui se paupérise.

écrivait en 1988 que l'intrusion de l'informatique dans les rapports de production risquait de « faire glisser la classe ouvrière entière vers la précarité, la fluidité imposée, l'instabilité de l'emploi et la multiplication des formes de travail précaire ». Nous y sommes. Sous couvert d'innovation technologique en faveur de l'autonomie, la réinstaure le salaire à la pièce, qui avait prospéré au XIX siècle et qui consistait à rémunérer les ouvriers des manufactures à la pièce produite plutôt qu'au temps horaire. Retour au XIX siècle, donc, quand Marx écrivait qu'il s'agissait là de la forme la plus optimale du capitalisme, car elle précarise les travailleurs à qui l'on propose des prix toujours plus faibles pour chaque pièce, tout en maximisant les profits. Ce tâcheronnage à la pièce, comme au XIX siècle, est le sort actuel des livreurs et celui des 250 000 microtravailleurs liés, en France, à d'autres plateformes que ce projet oublie d'ailleurs la République du Printemps des peuples- puisque nous sommes de nouveau au XIX siècle désormais -avait interdit le recours au salaire à la pièce. Voici qu'il revient, en 2021, en se faisant passer pour une solution futuriste, innovante, enviable pour les travailleurs. Or l'« ubérisation » n'est pas le futur. C'est la destruction des conquis sociaux. Pour les écologistes, il n'existe pas de dignité au travail sans droits sociaux,

regrette à mon tour que le Gouvernement recoure aux ordonnances pour légiférer sur le dialogue social des plateformes numériques. Outre le fait que le Gouvernement organise, une fois de plus, le dessaisissement du Parlement,

pour les travailleuses et les travailleurs des plateformes, mais uniquement des plateformes de mobilité, comme les chauffeurs VTC et les livreurs de repas. Ces 50 000 travailleurs, qui ne disposent d'aucune garantie en matière de revenu minimum, de conditions de travail ou de protection sociale pourront donc élire des représentants, dont on peut se demander ce qu'ils pourront bien négocier. Ce texte vise à sécuriser le modèle économique des plateformes et à éviter le risque de requalification salariale devant le juge, en renforçant le critère d'indépendance. Cette position est en totale opposition- faut-il le rappeler ? -avec la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans des arrêts en date du 28 novembre 2018 et du 4 mars 2020, a reconnu respectivement la qualité de salarié à un livreur de la plateforme Take Eat Easy et à un chauffeur Uber. Ce texte ajoute une nouvelle pierre à l'édifice, en créant un cadre de dialogue social entre travailleurs et plateformes sans aborder la question de leur statut.

préconisait de clarifier le statut de ces travailleurs, en proposant plusieurs scénarios, parmi lesquels celui de la reconnaissance d'un statut de salarié. de loi se résume à une tentative maladroite de s'inspirer du modèle du salariat en matière de négociation collective, sans pour autant appliquer aux travailleurs les protections minimales garanties par le code du travail. En quelques années, les plateformes numériques se sont développées de manière rapide, révolutionnant nos manières de communiquer, de consommer et de travailler.

Le modèle économique des plateformes reste fragile. Il repose principalement sur la possibilité de mobiliser des travailleurs pour un coût social bien moindre que l'emploi de salariés.

Triste aveu d'un système économique qui précarise des milliers de travailleurs, sans pour autant atteindre la prospérité ! Ces constats appellent à une régulation des plateformes numériques

Cette solution aurait un triple mérite : clarifier juridiquement le statut de ces travailleurs au regard du droit du travail et de la protection sociale, améliorer leurs conditions de travail et leur rémunération et, enfin, reconnaître leur dépendance économique à l'égard des plateformes dans l'exercice de leur activité. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera contre ce projet de loi de ratification et d'habilitation. La parole

humour votre interrogation quant au fait que la gauche de l'hémicycle ne souhaiterait pas le dialogue social ... Soyons sérieux ! Je vous connais, je ne peux prendre cela autrement qu'avec humour, même si la situation est grave. Madame la ministre, vous n'êtes pas Waldeck-Rousseau qui, en 1884, a permis aux syndicats

collective- ou plutôt au « dialogue social » pour faire écho à l'intervention précédente -plutôt que d'en fixer le cadre dans la loi. En cela, l'ordonnance maintient la fragilité de la position des représentants des travailleurs affaiblit la possibilité de réelles avancées quant à l'amélioration de leurs conditions de travail et renonce surtout à la transposition d'un certain nombre de droits sociaux susceptibles de les protéger par la loi. Or l'instauration d'un dialogue social sans droits sociaux l'encadrant ne fait pas grand sens. Le rapport de force est, de fait, inégal, entre plateformes et représentants des travailleurs. Il le sera d'autant plus si nous renonçons à poser un cadre renforçant les capacités de négociation de ces derniers. À cet égard, le rôle des institutions publiques aurait dû être de contrebalancer ces inégalités en protégeant les travailleurs par l'instauration de droits, et non d'abandonner les travailleurs face aux plateformes.

Nous sommes destitués de notre rôle. Encore une fois, les travailleurs font les frais de l'éviction de la démocratie sociale et parlementaire. Nous demandons la suppression de cet article, dans l'attente d'une loi

Madame la rapporteure, vous avez dit que ces nouvelles formes de travail avaient finalement permis

inadmissible ! Madame Puissat, j'aurais aimé vous entendre sur le fait que ce texte va clairement contribuer à créer un tiers-statut, alors que vous y étiez-

Lubin. Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2021 prévoyant des mesures dérogatoires en matière de représentativité des organisations de travailleurs, notamment un seuil de 5 % de suffrages exprimés pour le premier scrutin,

présenter l'amendement n° 22. L'article 2 du présent projet de loi organise le dessaisissement du Parlement, en habilitant une nouvelle fois le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l'instauration d'un cadre de dialogue social au niveau des plateformes.

à l'ARPE, puisque cette institution n'aura pour mission que d'organiser le dialogue et les élections sans que rien soit prévu pour qu'elle puisse intervenir en cas d'abus. Il semblerait que nous soyons ainsi devant une sorte de coquille vide. Nous dessaisissons le Parlement de son rôle et, dans la pure tradition néolibérale, nous transformons les organismes et établissements publics en agences d'organisation du marché, en laissant les travailleurs démunis face à leur hiérarchie de fait.

suppression de l'article 2. On ne peut pas faire l'économie d'un projet de loi et d'une discussion démocratique, sociale et parlementaire sur l'ensemble des droits sociaux des travailleurs, lorsqu'on

concertations. Il est clair que certains sujets seront incontournables, comme la détermination d'un revenu minimal d'activité, la sécurisation des parcours professionnels ou encore l'amélioration des conditions de travail. C'est d'ailleurs le sens de l'amendement n° 17 déposé par le Gouvernement, qui vise à préciser l'habilitation sur les thèmes qui pourront donner lieu à une négociation. Sur la méthode, l'intention du Gouvernement n'est pas d'empêcher le débat parlementaire, comme en atteste l'examen de ce projet de loi. Je le redis, je me tiens à la disposition du Parlement pour l'informer de manière régulière de l'avancée des travaux sur les projets d'ordonnances.

propose de rétablir l'habilitation à fixer par ordonnance les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire au niveau du secteur d'activité. Avant d'arrêter d'arrêter définitivement les différents thèmes possibles de négociation, il est nécessaire de pouvoir achever la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Pour autant, je partage avec vous le constat qu'il est important que la négociation sectorielle puisse traiter certains sujets centraux. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 17 propose de compléter l'habilitation pour préciser les thèmes qui pourront être traités par ce dialogue social entre les représentants des travailleurs et des plateformes : il s'agit notamment de la détermination des revenus des travailleurs, du développement des compétences professionnelles, la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs et des mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels, auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. Je crois, madame la rapporteure, que nous sommes toutes deux attachées à ce que ces sujets essentiels soient traités dans le dialogue social.

en sorte que le travailleur puisse choisir librement son itinéraire. Il n'est donc pas question de contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, comme vous le soutenez, mais d'en tirer toutes les conséquences pour s'assurer que les plateformes respectent bien les règles. Si elles ne le faisaient pas,

Le prix de la prestation constitue l'élément central de la négociation attendue, car c'est de celui-ci que découle, pour les travailleurs, la possibilité de percevoir un revenu décent et de financer, leurs cotisations sociales, leur protection sociale obligatoire et complémentaire. sociales, leur protection sociale obligatoire et complémentaire. Cette dernière doit être exclue du champ du fameux dialogue social, aussi bien à l'échelle de la plateforme que du secteur, et ce pour les raisons suivantes : cela reviendrait à créer un tiers-statut comportant des droits inférieurs à ceux des salariés, mais supérieurs à ceux des autres indépendants serait à l'origine d'une dépendance sociale, inacceptable selon nous, pour des travailleurs dits « indépendants », serait source d'une inégalité de traitement entre les travailleurs exerçant en nom propre et ceux qui travaillent pour les plateformes,

14. Par cohérence avec notre opposition de principe à la création d'un tiers-statut, nous souhaitons la suppression de cet article, introduit par Mme la rapporteure, car il participe de cette logique, et ce d'autant plus que la protection des travailleurs des plateformes y est renvoyée au dialogue social. Pour notre part, nous soutenons depuis plusieurs années la reconnaissance du salariat pour ces travailleurs et nous souhaitions instaurer dans ce projet de loi une présomption réfragable de relation de travail pour les travailleurs ayant recours à des plateformes. Malheureusement, notre amendement a été déclaré irrecevable dès son dépôt en commission, en application de l'article 45 de la Constitution. La parole est à Mme la ministre,

C'est en ce sens que nous avons rédigé cet article 3, avec un certain nombre de paramètres qui devraient quand même correspondre aux attentes des uns et des autres, puisque nous évoquons la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels. Je mets aux voix les amendements

Le scrutin est clos.

Pour dégager un salaire minimum, les études montrent qu'un livreur doit travailler de 14 heures à 15 heures par jour. La fluctuation des tarifs, leur imposition par la plateforme, l'augmentation des commissions

Nous devons préserver les droits et instituer une négociation sociale plus juste qui tende à contrebalancer l'inégalité des rapports de force. Pour ce faire, il faut qu'un tarif minimum égal au SMIC horaire soit institué, avec la garantie que la négociation autour du prix de prestation parte de ce tarif

inférieur au SMIC horaire. La question du prix est une préoccupation partagée par la commission, mais cette référence n'est pas appropriée dans le cadre d'une tarification à la prestation. En outre, il faut rappeler que le prix de la prestation n'est pas équivalent au revenu des travailleurs concernés, lequel dépend aussi de la commission prélevée par la plateforme et des charges acquittées par eux. Quel est l'avis du

Selon les études disponibles, il y a quinze fois plus de risques d'accident dans le métier de livreur chez Deliveroo que dans un métier de livraison classique. N'oublions

minute trente pour savoir s'ils acceptent une course, qu'ils doivent livrer au plus vite, faute de quoi la plateforme peut les déconnecter. La prévention des risques professionnels fait pourtant l'objet d'un cadre juridique très clair dans le code du travail. La préservation de la santé des travailleurs est un impératif et un droit fondamental. Nous ne pouvons plus laisser les plateformes mettre leurs travailleurs en danger sans encourir aucune responsabilité. L'amendement vise ainsi à renforcer la protection des travailleurs de plateforme contre les risques professionnels en insérant une référence claire aux dispositions du code du travail,

une préoccupation de la commission. Du reste, nous l'avons inscrite à l'article 3 dans le socle des négociations obligatoires qui devront avoir lieu au niveau sectoriel. Vous précisez dans votre amendement que ces négociations devront tenir compte des dispositions du code du travail sur la surveillance de la santé des travailleurs par les services de santé au travail. Or la loi du 2 août 2021

du Gouvernement ? Je confirme les propos de Mme la rapporteure. La loi Santé au travail du 2 août dernier prévoit en effet que les travailleurs indépendants peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix. Ils bénéficient alors d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Par ailleurs, ce sujet de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail

Instaurer un dialogue social sans droits sociaux revient à légiférer sur l'encadrement d'une coquille vide, ce qui ne pourra se faire qu'au détriment des travailleurs. Un certain nombre de droits sociaux de base manquent pour servir de cadre à ce fameux dialogue social. Il n'y a pas de garantie d'un tarif ou d'un revenu minimum, d'une durée maximale de travail, d'un encadrement des heures de repos, de congés payés, d'indemnités de licenciement, de droit de retrait. Sur quoi voulez-vous que les salariés discutent et négocient si aucune référence n'est faite à ces droits inscrits dans le code du travail ? Cet amendement vise donc à donner du contenu au dialogue social en ramenant ces ordonnances à des références claires au code du travail.

que nous protégerons les travailleurs et leur autonomie. que la commission a prévu que, dans ce cas, les organisations représentatives dans chaque secteur doivent négocier tous les ans sur la fixation du prix, et tous les deux ans sur le développement des compétences professionnelles et sur la prévention des risques professionnels.

d'avoir travaillé sur un texte de loi qui essaie d'offrir quelques bribes de protection sociale à des travailleurs précaires,

Je constate que nos positions n'ont pas totalement convergé, mais je pense que nous avons montré collectivement notre souhait de faire progresser les droits des travailleurs des plateformes en privilégiant la voie d'un dialogue social structuré et équilibré, qui permette aux travailleurs concernés de disposer d'un moyen de se faire entendre. Je voudrais rassurer M. le sénateur Savoldelli, ... Ça va être dur ! ... le ministère des transports est bien associé à ces travaux. S'agissant de la santé au travail, je vous précise qu'il s'agit d'une prérogative du ministère du travail.